La séance est ouverte.. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

et en application de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, M. le Premier ministre, par lettre en date du 24 janvier 2017, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission du Sénat compétente en matière d'environnement sur le projet de nomination de M. Philippe Martin aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. Cette demande d'avis a été transmise à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Acte est donné de cette communication. M. le Premier ministre a demandé à M. le Président du Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d'un sénateur appelé à siéger au sein de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. La commission de la culture a été invitée à présenter un candidat. La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de réunion d'une commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à cette commission mixte paritaire. Cette liste a été publiée conformément à l'article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n'est faite dans le délai d'une L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, avec le projet de loi qui est soumis à votre approbation la liaison ferroviaire Lyon-Turin va franchir une étape décisive vers sa réalisation. vers sa réalisation. Il a en effet pour objet d'autoriser l'approbation de l'accord du 24 février 2015 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Cet accord intergouvernemental marque la dernière étape de ce grand projet franco-italien et européen, né il y a déjà plus de vingt-cinq ans. Il fait suite à deux précédents accords intergouvernementaux : pour la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire permettant la création d'un promoteur public, signé en 2001 ; l'accord intergouvernemental pour définir les modalités de gestion du projet et instituer un nouveau promoteur public chargé de la conception, de la réalisation, puis de l'exploitation de la section transfrontalière, signé en 2012. Le présent accord, signé le 24 février 2015, vient compléter les deux précédents et comprend trois volets volets : il permet le lancement des travaux définitifs de la section transfrontalière ; son protocole additionnel valide le coût du projet certifié et en précise les modalités de financement ; le règlement des contrats met en place des dispositions de lutte contre la criminalité organisée, afin de vérifier les règles de passation de marché et les entreprises éligibles. Les enjeux de la création du tunnel Lyon-Turin sont majeurs. Sur un plan économique, d'abord, cet accord répond à un objectif de rééquilibrage des flux. Il y a aujourd'hui un risque que le trafic de marchandises en provenance du Benelux et du Royaume-Uni à destination de l'Italie se déplace progressivement vers la Suisse et l'Autriche, qui se dotent d'infrastructures modernes répondant aux standards ferroviaires de demain le tunnel du Gothard, le plus long tunnel ferroviaire du monde, inauguré en juin 2016, et celui du Brenner, en construction. Le lancement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la ligne ferroviaire Lyon-Turin va permettre d'asseoir la position de la France au coeur des échanges économiques européens. Le tunnel transfrontalier renforcera la compétitivité de nos entreprises et bénéficiera à nos relations économiques avec l'Italie, qui est notre deuxième partenaire commercial, mais aussi à nos relations économiques avec le reste de l'Europe. Il s'agit d'ailleurs non pas seulement de relier Lyon et Turin, ni même Paris et Milan, mais aussi de rapprocher les grandes zones économiques des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Piémont et Lombardie, qui représentent 3,2 % du produit intérieur brut de l'Union européenne. Par ailleurs, les retombées économiques de la création du tunnel seront importantes grâce à une démarche de « grand chantier » qui stimulera l'emploi et la croissance de la région. L'exploitation, l'entretien et le renouvellement de la nouvelle ligne ferroviaire, le renforcement de l'attractivité des territoires sont autant d'atouts pour la création d'emplois. La liaison Lyon-Turin est aussi la réalisation d'une grande infrastructure européenne, pleinement inscrite dans le corridor transeuropéen méditerranéen reliant la péninsule ibérique à la Slovénie et la Hongrie, qui fera de la France un centre de gravité de l'Europe, à un moment où le trafic entre l'Espagne et l'Italie augmente. enjeu majeur, également, sur le plan de l'environnement. Chaque année, ce sont en effet plus de 2,7 millions de poids lourds qui traversent nos vallées alpines et notre littoral. Ces véhicules empruntent des routes où le trafic de transit pose de graves problèmes, qu'il s'agisse de zones urbanisées et congestionnées- je pense notamment à l'autoroute A8 autour de Nice -, ou encore de zones très sensibles du point de vue environnemental. Les vallées de l'Arve et de la Maurienne sont particulièrement affectées par la pollution, comme nous l'avons vu ces dernières semaines Nous devons donc absolument favoriser le passage du transport de marchandises de la route vers le rail en facilitant le report modal. Le transport routier est dominant, mais cela ne peut pas durer. La majorité du trafic de marchandises qui emprunte les tunnels routiers des Alpes franco-italiennes parcourt des trajets de plus de 500 kilomètres et entre ainsi pleinement dans le domaine de pertinence du mode ferroviaire. Nous croyons à l'avenir du transport ferroviaire, en particulier pour le fret. pour le fret. Lors de la signature de la convention alpine en 1991, mais aussi plus récemment lors de la COP21, nous nous sommes engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le réchauffement climatique. Le tunnel Lyon-Turin est un élément important pour le respect de ces engagements, car il permettra au ferroviaire d'assurer plus de 40 % des échanges de marchandises dans la zone, à l'horizon 2035, contre 8,8 % en 2015, soit un report estimé à 700 000 poids lourds vers le rail. En ce qui concerne le transport de personnes, la création du tunnel Lyon-Turin améliorera la compétitivité du train par rapport à l'avion en termes de facilité d'accès et de rapidité. Le report modal permet également de renforcer la sécurité des transports dans cette zone transalpine. dans cette zone transalpine. Nous avons en mémoire les incendies mortels qui ont eu lieu dans les tunnels routiers des Alpes franco-italiennes en 1999 et 2005, et l'éboulement rocheux sur l'autoroute A8 en 2006. Les infrastructures ferroviaires existantes, notamment celle du Montcenis, qui date de 1871, ne peuvent pas offrir des services performants répondant aux besoins actuels du trafic. Une modernisation de ces infrastructures est donc indispensable au regard des flux de marchandises et d'usagers Qu'en est-il de la question du coût et du financement de ce projet ? Le protocole additionnel de l'accord soumis à votre approbation valide le coût certifié global du projet à 8,3 milliards d'euros en valeur 2012. Signe de son importance pour l'Europe, le projet bénéficie d'une subvention de 813,8 millions d'euros de l'Union européenne, au titre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, pour la période 2014-2019. octroyée pour la section transfrontalière, correspond aux taux maximaux possibles de cofinancement par l'Union européenne. Il reste ainsi pour la section transfrontalière 35 % à la charge de l'Italie et 25 % à la charge de la France. Avec Avec le maintien par l'Union européenne de sa participation à hauteur de 40 % au-delà de 2019, la contribution de la France s'élèvera à 2,21 milliards d'euros valeur 2012, soit 2,48 milliards d'euros courants. Ce financement ne pèsera pas exclusivement sur le budget de l'État ; on aura également recours aux crédits du Fonds de développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin, le FDPITMA. La part française des premiers travaux à la réalisation du tunnel de base sera financée en 2017 l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFITF. C'est tout à fait essentiel, et nous ne pouvions pas laisser passer ces financements européens. Très bien ! Nous nous sommes battus pour que le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe soit renforcé et doté de montants très importants dans la programmation européenne 2014-2020

25 % du financement de cette infrastructure, permettra à ce projet de voir le jour. Dernier point essentiel de cet accord l'instauration d'un règlement des contrats qui décline les dispositions de lutte contre les infiltrations mafieuses, prévues dans le droit italien et compatibles avec le droit de l'Union européenne. Ce règlement des contrats, d'une extrême rigueur, instaure une structure binationale inédite chargée d'écarter toute entreprise qui présenterait des liens avec la criminalité organisée. Son application sera contrôlée par un préfet français désigné par le Gouvernement, qui validera les refus d'inscription d'entreprises françaises sur la liste blanche. Une inscription sur cette liste blanche sera nécessaire pour toute entreprise souhaitant travailler sur le chantier de la partie centrale de la ligne. Cette inscription se fera selon des critères prenant en compte certaines condamnations pénales précisées dans le règlement, les infractions prévues dans le droit pénal français ou italien, mais également toute situation conduisant à suspecter que l'entreprise est contrôlée ou influencée par une organisation criminelle de type mafieux. En Italie, le Sénat et la Chambre des députés ont déjà donné leur aval à la ligne Lyon-Turin, respectivement le 16 novembre et le 20 décembre 2016. Le Président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, a promulgué la loi le 12 janvier 2017, finalisant ainsi la procédure de ratification en Italie. La France doit désormais faire de même. Le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin est en effet un projet d'avenir

dans la lutte contre le changement climatique. Il s'inscrit dans une dynamique de coopération et de cohésion nécessaire pour relancer le projet européen. Enfin, il est un acte de foi dans la coopération franco-italienne, dans le rapprochement entre nos pays et nos économies, et dans le projet européen lui-même. Nous avons obtenu, je le redis, une prise en charge majeure par l'Union européenne, dans le cadre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ce qui était essentiel à la réussite de ce projet. Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité. C'est pourquoi le Gouvernement a tout mis en oeuvre pour que nous répondions dans les délais à chacun des appels à projets et que nous soyons en mesure, avec nos partenaires italiens, de bénéficier pleinement des soutiens européens. La ratification de cet accord est donc nécessaire pour qu'aboutisse ce grand projet de nature à renforcer

et au tunnel ferroviaire du Fréjus, situé à plus de 1 300 mètres d'altitude, une ligne de plaine, plus compétitive et répondant aux standards internationaux.

entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse-Bussoleno, sera réalisée par le promoteur public, la société TELT- Tunnel Euralpin Lyon-Turin -, entre 2017 et 2029.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

fixe le coût certifié de la section transfrontalière à un peu plus de 8 milliards d'euros. La Commission européenne a attribué à ce chantier une subvention d'environ 810 millions d'euros, pour la période 2014-2019- nous espérons que l'Europe perdurera au titre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit une prise en charge des travaux à hauteur de 40 %, le taux maximal. La participation financière de la France s'élève à un peu plus de 2 milliards d'euros, soit 25 % du coût total du projet. Il importe de garantir la pérennité du financement par la France de 200 millions d'euros chaque année,

dans les contrats conclus par le promoteur public TELT, qui reprend la législation italienne en la matière. Je rappelle que, si le droit italien permet d'inscrire une entreprise sur une liste blanche

dit -, sera chargée de vérifier les motifs d'exclusion des contrats passés par TELT. Le préfet français effectuera ces contrôles sur les entreprises françaises sans disposer de moyens propres dédiés.

Enfin, récapitulons les enjeux de cette section ferroviaire transfrontalière, qui sont bien connus de tous. Tout d'abord, je veux évoquer le report modal du fret et des voyageurs de la route vers le rail et la sécurisation des transports. Actuellement, les flux routiers représentent 90 % des échanges de fret entre la France et l'Italie, et 2,5 millions de poids lourds traversent chaque année le massif alpin. La part modale du fer n'a cessé de diminuer.

La France s'est engagée en signant la convention alpine de 1991. Le train, quatre à cinq fois moins polluant qu'un transport routier, permettra la réduction des émissions de polluants, alors que la fréquence et la durée des pics de pollution sont en augmentation dans les Alpes. Enfin, la section transfrontalière

Il devrait permettre à terme un rééquilibrage géostratégique des flux économiques, en favorisant les échanges entre la France et l'Italie- notre deuxième partenaire en termes d'échanges commerciaux

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, près de trois millions de poids lourds passent par la frontière franco-italienne chaque année, soit 7 500 poids lourds par jour. En augmentation constante depuis quarante ans, le trafic se concentre sur trois axes majeurs, conduisant à une saturation des vallées alpines et de Vintimille, et parfois à des accidents majeurs. Nous gardons tous en mémoire l'incendie l'incendie dans le tunnel du Mont-Blanc en 1999 ou celui du tunnel de Fréjus en 2005. Rappelons également que la Savoie est aujourd'hui le département le plus pollué de France. Face à ces défis, il est impératif de permettre le report modal de la route vers le rail. Depuis 1970, la part modale est passée en France de 78 % à moins de 10 % pour le train et, à l'inverse, de 22 % à 90 % pour la route. La ligne ferroviaire historique passant par le Montcenis et le goulet d'étranglement de Saint-Jean-de-Maurienne est totalement saturée. Elle a atteint ses limites à la fin des années quatre-vingt-dix avec un tonnage de fret de plus de dix millions de tonnes par an. Les mesures mises en oeuvre pour tenter de la désengorger, comme l'ouverture du faisceau de Saint-Avre, se sont révélées largement insuffisantes. De la même manière, à défaut des deux tunnels sous les massifs de Chartreuse et de Belledonne, il est à craindre que des millions de tonnes de fret se déversent sur Chambéry, Aix-les-Bains ou le long du lac du Bourget, perturbant encore un peu plus un secteur ferroviaire dégradé pour les usagers.

Le tronçon alpin transfrontalier participera à la mise en place du corridor souhaité par l'Union européenne entre l'Espagne et l'Europe orientale. Ce projet s'inscrit donc dans une dynamique européenne favorisant à la fois le développement des transports et la protection environnementale des Alpes. La ligne Lyon-Turin doit ainsi constituer un investissement socialement et écologiquement utile répondant à plusieurs enjeux. Pour les voyageurs, ce projet entraînera une réduction significative du temps de trajet Lyon-Turin. Le report modal avec une ligne principalement dédiée au fret qui devrait représenter 85 % du trafic permettra également de soulager les axes routiers surchargés. En matière d'emplois, on estime à 3 000 le nombre de créations directes de postes dans la vallée de la Maurienne, et à 300 les emplois pérennes liés à l'exploitation du tunnel. Enfin, ce projet sera déterminant dans la lutte contre les pollutions et les nuisances locales. En outre, il ouvrira des possibilités nouvelles pour des cadencements et des TER « grande vitesse » directs entre Lyon et Grenoble, Chambéry et Annecy, ainsi qu'une amélioration des dessertes locales grâce à la libération de la ligne historique.

de promouvoir des transports rapides et moins polluants et de répondre aux besoins de mobilité des populations locales et des voyageurs.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au-delà de leur participation active dans la construction européenne, la France et l'Italie ont su préserver des relations bilatérales fortes. La liaison ferroviaire Lyon-Turin, comme bien d'autres projets de grande ampleur, constitue la vitrine d'une Europe unie capable d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Après une genèse quelque peu laborieuse, l'accord du 24 février 2015, son protocole additionnel du 8 mars 2016 et le règlement des contrats annexé soumis à l'approbation du Parlement confirment l'engagement définitif des travaux de la section transfrontalière de la ligne ferroviaire. Ils définissent les conditions de leur réalisation. La certification du coût prévisionnel du projet par un tiers extérieur était une condition de la signature par la France de cet accord. C'est chose faite ; selon les hypothèses retenues, il représentera 8,3 milliards d'euros en valeur 2012 ou 9,6 milliards d'euros courants, la France intervenant à hauteur de 25 %, soit un peu plus de 200 millions d'euros par an entre 2017 et 2029. Depuis l'accord de Rome signé le 30 janvier 2012, la participation financière de l'Union européenne à hauteur de 40 % a été confirmée, comme nous l'espérions, puisque la nouvelle ligne ferroviaire constitue une partie intégrante du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen. Mes chers collègues, les enjeux sont de taille, et je rappellerai brièvement l'utilité sociale, économique et écologique de ce projet pour nos deux pays. Premièrement, il présente des avantages en matière d'aménagement du territoire en garantissant une desserte plus efficace des territoires de l'arc que ce soit pour le transport des personnes ou des marchandises. C'est l'occasion tant attendue de relancer la politique ferroviaire du fret, en régression dans notre pays malgré les besoins réels de nos entreprises. Deuxièmement, la nouvelle liaison ferroviaire facilitera les échanges commerciaux et devrait être bénéfique pour l'économie locale. En effet, l'axe routier est saturé et la ligne historique pose de graves problèmes de sécurité et de fiabilité en raison de son obsolescence et des particularités géographiques que l'on connaît. Troisièmement, et ce n'est pas pour autant le point le moins important, on peut citer le report sur le mode ferroviaire d'une partie des 3 millions de poids lourds traversant tous les ans le massif alpin. Le projet participera, dès lors, à la mise en oeuvre de la convention alpine signée en en 1991 et aux objectifs ambitieux de la France et de l'Union européenne en termes de réduction de gaz à effet de serre : il permettra aux habitants des zones concernées de respirer un air de meilleure qualité. Comme vous l'aurez compris, le groupe du RDSE soutient la réalisation

Toutefois, c'est bien l'aberration économique et financière que représente la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre Lyon et Turin qui nous interroge. C'est parti ... Si le désengorgement des axes routiers était bien l'objectif environnemental de ce projet en 1991, les prévisions qui ont présidé à son lancement se sont révélées être très largement surévaluées. Alors qu'il était initialement prévu 19 millions de passagers après la mise en service de cette ligne, Réseau ferré de France n'en prévoyait plus que 4,05 millions est la même pour le fret dans les Alpes du Nord : alors qu'il était prévu une explosion des échanges, le transport de marchandises, du fait de la désindustrialisation, est passé de 35 millions de tonnes entre 1994 et 1998 à 22 millions de tonnes aujourd'hui. Au regard de la nouvelle donne du trafic, si ce projet avait un sens au début des années quatre-vingt-dix, c'est bien son utilité aujourd'hui, en 2017 et dans les années à venir, que nous contestons, d'autant que l'on sait que la voie ferroviaire existante est utilisée à moins de 20 % de sa capacité. Alors que de nombreuses lignes sont encore en voie unique, le doublement des voies et leur sécurisation pourraient permettre d'absorber une grande partie du trafic routier dans la région au travers d'une hausse de la fréquence. Il existe donc des solutions alternatives valables pour lutter contre la pollution et les conséquences du trafic routier sur l'environnement, et ce à moindre coût. C'est en effet justement l'explosion des coûts du projet qui nous interpelle, nous, mais pas seulement. En 2012, la Direction du trésor a évalué le projet global à 26,1 milliards d'euros, contre 2,1 milliards d'euros initialement prévus. Pour la seule section transfrontalière, le coût est quant à lui estimé à 8,3 milliards d'euros, contre 4,5 milliards d'euros initialement. Selon la Cour des comptes, le financement du projet n'était toujours pas précisé en 2016, condition pourtant exigée par l'accord franco-italien du 30 janvier 2012 pour le lancement des travaux. Pis encore, dès 1998, le Conseil général des ponts et chaussées mettait en garde contre la faible rentabilité socio-économique de ce projet et l'absence de financement. Devant des prévisions erronées et un coût qui explose, il apparaît nécessaire, conformément à l'avis du groupe de travail sur le financement des infrastructures de transport de la commission des finances, que le Commissariat général à l'investissement mène une contre-expertise indépendante de l'évaluation socio-économique pour des projets supérieurs à 100 millions d'euros et donc pour la liaison Lyon-Turin. Dans un contexte de raréfaction de l'argent public, l'État français, les collectivités territoriales et le contribuable sont-ils en mesure de supporter une telle charge ? N'est-ce pas l'ensemble du réseau ferré français qui nécessite aujourd'hui un investissement massif ? Le président de la SNCF a lui-même reconnu que le projet Lyon-Turin serait « autant d'argent en moins pour moderniser le réseau ferroviaire existant ». Il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement aux grands travaux, mais de poser la question des choix que nous opérons en matière d'aménagement du territoire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, après les ratifications à des majorités massives des accords précédents conclus avec l'Italie sur le même projet, le 29 janvier 2001 et le 30 janvier 2012, et le débat que nous avons eu au sein de la commission des affaires étrangères du Sénat, l'issue positive du débat ne fait aucun doute,

où une bonne partie de la France tousse, où la pollution nous rend malades- permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les vallées alpines -, je veux rappeler toute l'importance de la modernisation de cette traversée des Alpes, ainsi que l'intérêt écologique et environnemental du projet.

Les détracteurs du projet se gardent cependant bien de préciser que, pour réduire l'usage de leurs routes par les poids lourds, les Suisses ont largement subventionné l'exploitation fret de leurs lignes ferroviaires historiques, attirant ainsi vers leur pays, même si tel n'était pas leur projet, un trafic qui avait historiquement emprunté l'itinéraire alpin franco-italien.

sur l'exploitation de leurs lignes historiques devenues, de longue date, non compétitives. Enfin, on ne fera pas l'injure aux détracteurs du projet de croire qu'ils n'ont pas compris que la Suisse se dispenserait de la lourde dépense correspondant à la construction de tunnels de base, à leur charge exclusive, si elle ne considérait pas qu'il était temps pour elle de supprimer les pentes d'accès et de réduire l'altitude des tunnels de ses lignes historiques. Très bien ! En tout état de cause, une offre de transport ferroviaire pour le fret présente, en plus de ses conséquences écologiques particulièrement bénéfiques, le triple intérêt de réduire les consommations d'énergie, d'alléger les coûts de franchissement d'un massif comme les Alpes et d'assurer des gains de temps significatifs. Tous ces éléments constituent de fortes incitations au report de la route au rail du transport des marchandises, qui constitue un avantage environnemental capital.

il est d'autant plus indispensable et urgent de mener à bien le projet ferroviaire Lyon-Turin si l'on veut permettre à la France et à l'Italie : de rester compétitives avec leur unique liaison de franchissement est-ouest des Alpes ; de respecter à leur tour les engagements de report modal auxquels elles ont souscrit en signant la convention alpine ; de lutter contre les pollutions liées au trafic de poids lourds dans les vallées alpines- le bilan carbone du projet apporte de précieuses indications sur la réduction des émissions nocives tant pour les humains que pour l'environnement

Les motivations essentiellement franco-italiennes ne sont pas les seules justifications de la réalisation de la liaison Lyon-Turin. En effet, maillon clé du corridor méditerranéen du réseau central européen arrêté en 2011 et 2013 à Bruxelles, cette liaison est pour l'Union européenne la condition du rééquilibrage du continent entre l'Europe anglo-saxonne et l'Europe latine, et plus largement l'Europe du Sud, de la péninsule ibérique au centre de l'Europe. Pour mémoire, il faut rappeler que les échanges économiques concernés par les traversées du massif alpin s'élèvent annuellement à 105 milliards d'euros pour les traversées nord-sud et à 70 milliards d'euros pour les traversées est-ouest.

atteint aujourd'hui 150 millions de tonnes, avec une progression du trafic poids lourds de 1 % de 2009 à 2015 et de 6 % en 2015 et 2016.

un enjeu de sécurité. Il importe de rappeler que le tunnel historique est un tunnel monotube d'environ 13 kilomètres réalisé il y a plus d'un siècle et demi sur l'initiative de Cavour, avant que la Savoie soit rattachée à la France.

La semaine dernière, un grand quotidien national présentait la stratégie économique de la Chine et sa volonté de recréer une nouvelle route de la soie, avec une liaison ferroviaire de l'est de la Chine à l'Ouest européen qui, depuis 2014, permet déjà à un convoi de conteneurs de partir chaque jour de l'Allemagne pour rejoindre la Chine.

illustre à quel point l'infrastructure du Lyon-Turin, de par sa situation au coeur du corridor sud-européen, est une opportunité pour la France de ne pas se disqualifier au sud de l'Europe, comme malheureusement elle l'a fait sur sa façade maritime au nord. Oui, le Lyon-Turin est l'infrastructure des défis de demain.

pour la quatrième fois, nous sommes amenés à approuver une convention internationale entre la France et l'Italie portant sur la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Cet accord vise à engager le lancement enfin effectif des travaux de la section transfrontalière de cette nouvelle ligne ferroviaire. Il est complété par un protocole additionnel qui fixe, quant à lui, le coût certifié du projet et ses modalités de financement. Nous verrons si tout cela clôt le dossier, lequel a connu, nous le savons, de nombreuses difficultés. Au-delà de son caractère technique, l'accord confirme la volonté des deux pays de réaliser cet ambitieux projet d'infrastructure de dimension européenne dont ils peuvent espérer de nombreuses retombées. Comme l'a rappelé excellemment le rapporteur Yves Pozzo di Borgo, ce projet structurant, qui entre dans sa phase de réalisation, représente un intérêt économique majeur pour les deux pays concernés, mais aussi pour l'Europe. L'objectif de la ligne Lyon-Turin est de réduire sensiblement le temps de trajet entre Paris et Milan, de permettre un report modal du trafic de marchandises traversant les Alpes franco-italiennes et d'améliorer les liaisons entre les vallées et les grandes agglomérations alpines de France et d'Italie, en contribuant à effacer la barrière alpine. l'intérêt principal de cette ligne est d'organiser le report modal du trafic de marchandises de la route vers le ferroviaire dans les Alpes, qui ne peut se faire avec la ligne ferroviaire existante. En effet, 85 % des échanges passant par la frontière franco-italienne sont aujourd'hui routiers. Cette ligne est donc un facteur de développement du fret ferroviaire comme des échanges commerciaux entre la France et l'Italie. Au titre des bénéfices environnementaux du projet, on peut relever qu'il participe d'une politique de développement durable et de protection des Alpes. Le report modal sur la ligne ferroviaire diminuera l'ensemble des émissions de gaz nocifs liées au trafic routier et participera à la réduction des nuisances sonores. Je voudrais également souligner la dimension européenne de cette infrastructure. La ligne ferroviaire Lyon-Turin est un élément de l'Europe des transports puisqu'elle fait partie du réseau transeuropéen des transports, qui est un vaste schéma de connexions entre les différentes parties de l'Europe au moyen de dix corridors. En tant qu'axe de franchissement des Alpes, elle constitue un élément clé du corridor transeuropéen méditerranéen reliant la péninsule ibérique à l'Europe centrale et orientale, en faisant communiquer des bassins économiques majeurs en Europe. la liaison Lyon-Turin est un élément de compétitivité et d'emploi, car elle est un facteur de développement des échanges commerciaux et économiques entre les régions qu'elle dessert et traverse. Cela explique d'ailleurs pourquoi l'Europe finance une bonne partie du projet, à hauteur de 40 %.

du projet. Ce débat intervient également après plusieurs semaines de pollution persistante dans les vallées alpines, la vallée de l'Arve et la cluse de Chambéry notamment. La part du trafic routier dans ce phénomène n'est niée par personne.

sauf à admettre le déclin des ports français au bénéfice de l'hinterland des ports allemands et de l'Europe du nord, qui ne peuvent que se renforcer au travers des liaisons ferroviaires réalisées sur les axes nord-sud, entre la Suisse et l'Italie par exemple, ou entre l'Autriche et l'Italie.

La séance est reprise. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été publiée conformément à l'article 12 du règlement. Je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire : Titulaires : MM. Jean-Claude Lenoir, Ladislas Poniatowski, Daniel Laurent, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Roland Courteau, Franck Montaugé et Jean-Pierre Bosino. Suppléants : M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Marc Daunis, Daniel Dubois, Joël Labbé, Mmes Élisabeth Lamure et Sophie Primas. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro, signé à Bruxelles le 19 mai 2016, qui est soumis à l'examen du Sénat, est important puisqu'il concourt à nos efforts de stabilisation des Balkans occidentaux. Après les adhésions à l'OTAN de la Slovénie en 2004, de la Croatie et de l'Albanie en 2009, celle du Monténégro sera un gage de stabilité pour cette région,

Notre pays a dans ce domaine une responsabilité particulière, liée à l'histoire et au rôle qui a été le sien dans les Balkans au cours des vingt dernières années, responsabilité qu'il assume aujourd'hui pleinement dans le cadre des processus de coopération régionale et de dialogue, le processus de Brdo-Brioni, d'une part, et de Berlin, d'autre part.

a signifié sa volonté de se rapprocher de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et d'en devenir membre. Il a été invité par les alliés, en décembre 2009, à rejoindre le plan d'action pour l'adhésion, qui donne le statut officiel de candidat et engage formellement le processus d'adhésion. Dans le cadre d'un dialogue étroit avec l'OTAN, le Monténégro a conduit de nombreuses réformes. Il a fait d'importants efforts en matière de modernisation des forces armées et de réforme du secteur de la sécurité et du renseignement, comme l'ont souligné plusieurs rapports de progrès de l'OTAN. L'effort de défense du pays a été porté à 1,7 % du PIB, légèrement en deçà de l'objectif de 2 % que se sont fixé les alliés lors du sommet du Pays de Galles en septembre 2014. Le Monténégro a également conduit des réformes dans le domaine de la justice, pour renforcer l'indépendance du système judiciaire, intensifier la lutte contre la criminalité organisée et la corruption et assurer l'État de droit. Ces progrès ont été salués lors des sommets de Lisbonne en 2010 et de Chicago en 2012. Le sommet du Pays de Galles de septembre 2014 a ouvert un dialogue renforcé avec le Monténégro en vue de permettre aux alliés de se prononcer, à la fin de l'année 2015, sur l'opportunité d'une adhésion à l'OTAN. Lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'OTAN des 1 et 2 décembre 2015, les alliés ont donc pris par consensus la décision d'inviter le Monténégro à engager d'ultimes pourparlers en vue de son adhésion. Cette démarche a abouti, le 19 mai 2016, à la signature par les États membres de l'OTAN du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro. Le Monténégro a alors obtenu le statut de pays invité et a pu ainsi participer au sommet de l'OTAN à Varsovie, en juillet 2016. La ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro permettra à ce pays de devenir le vingt-neuvième allié de l'OTAN. Vingt et un des vingt-huit membres de l'Alliance atlantique ont d'ores et déjà ratifié ce protocole. Pour la France, l'adhésion du Monténégro à l'OTAN sera bénéfique, car ce pays joue un rôle important dans la région des Balkans occidentaux. Le Monténégro a recouvré son indépendance, perdue après la Première Guerre mondiale, le 3 juin 2006, en se séparant pacifiquement, par référendum, de la communauté de Serbie-et-Monténégro. Son indépendance a été reconnue immédiatement par l'ensemble de la communauté internationale et, je veux y insister, le Monténégro n'est en litige territorial ou diplomatique avec aucun de ses voisins. Il est au contraire un élément moteur de la coopération régionale dans les Balkans. Malgré sa taille modeste, la contribution du Monténégro à la sécurité de l'Alliance sera réelle. Entre l'Albanie et la Croatie, ce pays assurera un géographique le long de l'Adriatique, qui a son importance stratégique en matière de défense collective. Ce point était particulièrement important pour nos alliés de la zone. Le Monténégro participe d'ores et déjà comme partenaire, à la mesure de ses moyens, à plusieurs opérations de stabilisation

Son adhésion s'inscrira donc dans la continuité de cet engagement. Concernant la politique de l'OTAN en matière d'élargissement, je tiens à rappeler que l'ouverture du processus d'adhésion au Monténégro s'est faite dans le cadre d'un accord plus large entre alliés sur le traitement des questions d'élargissement de l'OTAN. la France s'est assurée, en amont du sommet de Varsovie, que l'invitation faite au Monténégro ne serait pas le signal d'un élargissement non maîtrisé. Pour la France, l'adhésion du Monténégro n'ouvre en aucun cas la voie à une relance générale de la politique dite « de la porte ouverte Pour la France, l'élargissement de l'OTAN n'est aujourd'hui ni une priorité ni une fin en soi. Il ne peut s'envisager que dans la mesure où il renforce effectivement la sécurité de l'espace euro-atlantique et la crédibilité de la défense collective.

nous avons accepté de considérer les mérites propres du Monténégro, mais nous avons veillé à ce que soit parallèlement adoptée une série de conditions destinée à d'autres pays candidats, pour l'adhésion desquels il n'existe pas aujourd'hui de consensus. L'accord entre alliés sur ce point, dont les principes ont été repris dans le communiqué du sommet de Varsovie, Varsovie, précise bien que l'attribution d'un plan d'action pour l'adhésion reste une étape incontournable pour la Géorgie ; que c'est aux pays candidats de prendre les mesures nécessaires s'ils souhaitent avancer sur la voie de l'adhésion, et non aux alliés de renoncer aux conditions posées que les candidatures seront évaluées, en priorité, à l'aune de la capacité des candidats à assumer les responsabilités et les obligations liées au statut de membre et, en particulier, à contribuer à la sécurité de l'espace euro-atlantique. Rappelons-nous qu'au lendemain de la guerre froide, l'élargissement de l'OTAN a été un facteur de renforcement de la sécurité du continent européen. Une forte demande de stabilité et de sécurité émanait des ex-pays membres du pacte de Varsovie. Tout comme l'Union européenne, l'Alliance y a répondu en définissant des modalités d'accession flexibles. L'objectif était de contribuer à une vaste architecture de sécurité européenne, où les processus d'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne étaient perçus comme complémentaires, tout en étant clairement distincts. ans plus tard, nous continuons de refuser l'idée d'un partage de l'Europe en sphères d'influence, comme celle d'un droit de regard extérieur sur le processus d'adhésion. La dégradation durable de notre environnement stratégique a cependant conduit l'OTAN à reconsidérer les perspectives d'élargissement actuelles. Nos partenaires comprennent bien désormais que les candidats à l'adhésion doivent être considérés, en premier lieu, en fonction de leur capacité à contribuer à notre défense collective et de la capacité de l'OTAN à garantir leur sécurité. Voilà en résumé, mesdames, messieurs les sénateurs, les enjeux de la ratification de ce protocole.

Je vous invite donc à juger ce projet de loi pour ce qu'il est : un développement circonscrit au cas du Monténégro, dont l'adhésion à l'OTAN sera positive pour la stabilité des Balkans occidentaux.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, peu après son indépendance, recouvrée en 2006 après des années d'intégration dans l'ensemble yougoslave puis d'union avec la Serbie, le Monténégro a fait part de son souhait de rejoindre la communauté euro-atlantique, souhait également manifesté par sa candidature à l'Union européenne. Pour ce pays multiethnique et multiconfessionnel, qui se situe dans une zone de turbulences, il s'agit avant tout de garantir sa sécurité et sa stabilité. De fait, l'accession du Monténégro à l'Alliance atlantique s'inscrit dans la politique dite « de la porte ouverte » appliquée à l'égard des pays de l'est de l'Europe après la fin de la guerre froide, et dont l'objectif était d'abord politique il s'agissait d'oeuvrer à la stabilité de la zone euro-atlantique, en promouvant dans ces pays la paix, la liberté et la démocratie. Le Monténégro fait partie de la dernière vague d'élargissement de l'OTAN, lancée à l'occasion du sommet de Bucarest de 2008, et dont la mise en oeuvre, convenons-en, s'est avérée problématique. Si l'Albanie et la Croatie sont assez rapidement parvenues à l'adhésion, le Monténégro est aujourd'hui le seul pays parmi les autres candidats- yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie -à remplir les conditions pour devenir membre de l'OTAN. Certes, il ne s'agit pas d'idéaliser ce pays, qui a encore des progrès à accomplir, notamment en tant qu'État de droit et en matière de lutte contre la corruption. Le Monténégro n'en a pas moins franchi avec succès les différentes étapes du processus d'adhésion, depuis le plan d'action pour l'adhésion

D'un point de vue militaire, il faut l'admettre, sa contribution financière au budget de l'Alliance sera modeste. Néanmoins, ce pays compte augmenter son effort de défense dans les années à venir, tant pour renforcer les effectifs de ses forces armées que pour renouveler ses équipements militaires, ses priorités de modernisation étant définies en fonction des objectifs d'intégration à l'OTAN. En outre, le Monténégro prend activement part aux opérations extérieures, dans le cadre de l'OTAN, avec une contribution à l'opération en Afghanistan, ou dans celui de l'Union européenne, avec notamment une participation à l'opération Atalanta de lutte contre la piraterie. Il faut souligner à cet égard la sensibilité maritime que le Monténégro est susceptible d'apporter à l'Alliance atlantique, qui pourrait s'avérer utile pour le traitement des problématiques méditerranéennes, comme la question des migrants. Enfin, d'un point de vue stratégique, l'entrée du Monténégro dans l'OTAN permet d'établir une continuité dans la défense européenne sur la côte Adriatique, en complétant le chaînon manquant entre la Croatie et l'Albanie.

Si elle paraît ainsi pouvoir être justifiée par des raisons objectives, l'adhésion du Monténégro à l'OTAN n'en reste pas moins une question discutée, tant sur le plan interne que sur le plan international. Pour une partie de l'opinion publique monténégrine, marquée par les bombardements de l'OTAN contre la Serbie, cette adhésion ne va pas de soi. La question a même été l'un des mots d'ordre des manifestations organisées contre le pouvoir à l'automne 2015. Elle a également occupé une large place dans les débats qui ont précédé les élections législatives du 16 octobre 2016, qui se sont accompagnées d'une tentative de déstabilisation du pouvoir. Ces élections n'en ont pas moins été largement remportées par des formations favorables à l'accession à l'OTAN.

Plus que les intérêts économiques et les liens culturels liés à la présence d'une forte minorité slave qu'entretient la Russie dans ce pays, c'est surtout la perspective d'un nouvel élargissement de l'OTAN, dans un contexte de tensions exacerbées avec cette organisation qui explique la réaction russe. En effet, la Russie considère que l'expansion de l'OTAN constitue une menace directe pour sa sécurité. Selon la dernière version de la doctrine militaire russe, il s'agit même du premier danger militaire auquel la Russie est susceptible de faire face. Comme l'ont souligné nos excellents collègues Robert del Picchia, Josette Durrieu et Gaëtan Gorce dans leur rapport de 2015 sur les relations avec la Russie,

s'agissant du Monténégro, pays de 620 000 habitants qui, de surcroît, ne borde pas les frontières russes, cette réaction relève davantage d'une position de principe qu'elle ne traduit un réel enjeu stratégique. Après un débat approfondi, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s'est donc finalement prononcée pour la ratification du protocole d'adhésion du Monténégro à l'OTAN. en effet de ne pas décevoir les attentes d'un pays méritant, qui s'est résolument engagé dans cette voie et en a franchi avec succès les différentes étapes, de conforter un pôle de stabilité dans les Balkans au bénéfice des pays voisins,

à l'heure où l'OTAN et l'Europe sont fragilisées par les déclarations du nouveau président américain, de mettre à mal l'unité de l'OTAN en rejetant ce texte alors qu'une grande majorité d'États alliés

En revanche, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées considère que, après cette adhésion, qui, soulignons-le, n'est en aucune manière dirigée contre la Russie, un terme doit être mis à la dynamique d'élargissement de l'OTAN ; l'adhésion à l'Alliance atlantique de pays comme la Géorgie, l'Ukraine, la Serbie représente pour la Russie une ligne rouge. Il est à cet égard nécessaire de poursuivre les efforts de dialogue et de coopération avec la Russie dans le cadre du conseil OTAN-Russie, qui, après avoir suspendu ses activités du fait de la crise ukrainienne, a tenu trois réunions durant l'année 2016, ce qui est un signe encourageant.

Cette intégration s'inscrit dans la stratégie développée depuis 1999 par l'OTAN et consistant à s'étendre à l'est de l'Europe. L'adhésion du Monténégro n'est qu'une étape supplémentaire de cette politique expansionniste, dans la continuité de l'intégration de douze autres pays de l'Europe orientale, multipliant ainsi les initiatives conduisant à l'isolement de la Russie et les tentatives d'implantation de matériel militaire dans les pays frontaliers. Cette dynamique, entamée malgré les accords signés avec Mikhaïl Gorbatchev en 1990 puis avec Boris Eltsine en 1997, prend encore plus d'importance pour l'organisation atlantique maintenant que le pouvoir de Vladimir Poutine se renforce. Cette volonté d'isoler la Russie en renforçant les positions de l'OTAN sur le flanc oriental vise en réalité à revenir à une logique de guerre froide. Soutenir ce projet revient à prendre le risque de nous entraîner dans une spirale de tensions, de provocations et de course à l'armement. Cette stratégie est si dangereuse que le ministre allemand des affaires étrangères, Frank-Walter Stenmeier, s'inquiète d'un tel projet et a affirmé : « Celui qui croit augmenter le niveau de la sécurité avec des parades de chars sur le front est de l'Alliance se trompe. Force est de constater que l'OTAN est restée crispée sur une logique désuète d'affrontement Est-Ouest, alors que le monde est incontestablement devenu multipolaire. Après le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN et l'adoption du projet de loi autorisant la ratification du protocole de Paris sur l'OTAN, la France a renoncé à son indépendance sur la scène internationale et notre diplomatie s'est inscrite dans une vision atlantiste. Or la promotion d'idéaux de paix et de coopération internationale est inconciliable avec le soutien à une organisation qui impose à ses membres une course aux armements tout en se dédouanant des résolutions de paix de l'ONU. À l'heure où les États-Unis, qui dirigent l'OTAN et sont toujours dépositaires du traité de Washington, viennent d'élire un président souhaitant revenir sur l'article 5 du traité sur le principe d'assistance mutuelle face aux menaces, il est temps pour la France de retrouver une voix indépendante dans le concert des nations. Notre pays a vocation à défendre un monde multipolaire en s'appuyant sur ses valeurs de défense des droits de l'homme partout dans le monde et en agissant en faveur d'une coexistence pacifique entre les peuples. tant qu'organisation de paix et de sécurité mondiale, un rôle fondamental à jouer dans ce nouvel ordre international. Elle doit s'affirmer comme l'instance par excellence de médiation et de règlement des conflits internationaux, et la France doit agir en ce sens. Persuadés que la résolution des conflits doit s'appuyer sur la politique et les résolutions de l'ONU, convaincus que la politique de course à l'armement de l'OTAN ne peut que conduire à la multiplication des conflits,

du pacte de Varsovie. L'entrée en vigueur du protocole signé à Bruxelles avec le Monténégro le 19 mai dernier s'inscrit dans cette logique en ouvrant l'OTAN à un État des Balkans

Tout d'abord, le sommet du Pays de Galles de 2014 a souligné que, depuis 2009, le Monténégro avait progressé dans l'application du MAP, le plan d'action pour l'adhésion. Ensuite, le Monténégro participe déjà à une mission de l'OTAN en Afghanistan. En outre, si l'intérêt d'une adhésion à l'OTAN est seulement jugé selon la capacité du pays candidat à contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord, on ne peut pas occulter les aspects relatifs à l'État de droit ; or, sur ce point, quelques indicateurs, issus des négociations

celle-ci reposant, je le rappelle, sur des exigences fortes en matière d'État de droit et de lutte contre la criminalité organisée. toujours du point de vue du processus d'adhésion, j'ajoute qu'une majorité de la population monténégrine l'approuve. Depuis les dernières élections de 2016, la majorité du Parlement est constituée de partis favorables à l'adhésion du

Si le cas du Monténégro peut encore passer, nous savons qu'il en sera autrement pour d'autres candidats, en particulier la Géorgie, l'Ukraine et la Serbie. Ainsi, puisque dix-neuf des vingt-huit États membres de l'Alliance ont procédé à la ratification du protocole, la France ne peut pas envoyer un mauvais signal ; de plus, compte tenu des avancées

L'enjeu du projet de loi dont l'examen nous réunit ce matin consiste donc à affirmer l'ancrage démocratique, libéral, au sens premier du terme, et occidental de ce pays d'Europe orientale. Le Monténégro a réalisé en une décennie un travail important pour affirmer son autonomie et sa viabilité en tant que nation indépendante.

Cette opposition est d'ailleurs pleinement associée à la vie politique du pays dans un cadre institutionnel qui avance à grands pas vers les standards modernes de la démocratie. Dans cette région, cela doit être souligné. À cet égard, je rappelle que le Monténégro, qui a affirmé son souhait d'adhérer à l'Union européenne dès 2008 est officiellement entré en négociation avec l'Union européenne il y a un peu plus de quatre

de la maturité de l'État du Monténégro dans le concert européen, cette adhésion présenterait un double avantage. Pour l'OTAN, intégrer le Monténégro facilite le travail de stabilisation des tensions récurrentes dans les Balkans-

Pour le Monténégro, cette adhésion est un stimulus indéniable pour la modernisation de son outil de défense. Nous sommes ainsi confrontés à un accord clairement gagnant-gagnant. Cet accord est d'autant plus stratégique sur le plan de la pure géopolitique que l'adhésion du Monténégro permettrait d'assurer la continuité territoriale de l'Alliance sur la côte Adriatique, de l'Albanie à la Croatie, tout en ouvrant des capacités d'intervention pour l'Alliance au Kosovo, en Bosnie et en Serbie.

Nos conclusions nous amènent à considérer que l'OTAN ne saurait désormais s'étendre dans la région au-delà du Monténégro, sauf à constituer une provocation à l'égard de notre voisin russe, qui voit dans l'OTAN, aujourd'hui encore, une menace pour sa sécurité.

pour les relations transatlantiques et l'incertitude dans laquelle elles se trouvent. D'une part, les propos virulents tenus par Donald Trump contre le modèle européen, mais également contre l'OTAN nous obligent à nous interroger sur le futur positionnement stratégique des États-Unis. part, dans le contexte de tensions exacerbées que nous traversons, notamment pour ce qui touche aux relations entre l'Union européenne et la Russie, l'intégration du Monténégro au sein de l'OTAN est-elle pertinente et souhaitable ? la question des répercussions de cette adhésion et du message qu'elle tend à véhiculer se pose tout de même, surtout quand on sait que la Russie a qualifié cette intégration de « provocation » et que l'on connaît les relations étroites qu'elle entretient avec le Monténégro. Il ne faut évidemment pas fermer la porte à toute évolution positive pour le Monténégro, marqué aujourd'hui encore par la corruption et la criminalité organisée, et les partenariats existants à la fois avec l'OTAN au travers du partenariat pour la paix et avec l'Union européenne au travers du partenariat oriental poussent le pays à se réformer non seulement militairement, mais aussi du point de vue de l'État de droit et doivent, selon nous, être poursuivis et renforcés. c'est la stratégie de fond que sous-tend ce protocole qui appelle notre attention, dans la mesure où celui-ci vise à asseoir un peu plus la primauté de l'OTAN au détriment d'une défense européenne. S'il faut bien évidemment reconnaître que l'OTAN est l'une des seules coalitions internationales où les armées aient réussi à coopérer, l'expérience récente d'une divergence fondamentale d'intérêts entre ses différents membres soulève la question de la pertinence d'un élargissement. La défense de l'Union européenne est aujourd'hui clairement déléguée à l'OTAN. l'Union doit assumer les responsabilités incombant à un acteur politique et économique de son rang. Il ne peut revenir aux États-Unis ni de nous protéger contre l'éventualité tragique d'une guerre ni de présider aux choix européens en matière de défense. Dans le contexte géopolitique changeant et incertain dans lequel nous vivons, pouvons-nous encore faire l'économie d'une relance de la défense européenne ? Alors que le modèle européen est en proie à des déstabilisations de toute part, n'est-il pas temps de dépasser les déclarations d'intentions et d'avancer concrètement sur ce dossier ? Je n'ai de cesse de rappeler devant vous la nécessité que l'Europe soit un acteur politique stratégique autonome, mettant son influence au service du système de sécurité collective et de la prévention ou la résolution des conflits. Pour ce faire, nous devons impérativement actualiser la stratégie européenne de sécurité, encourager un consensus politique en matière de défense et poursuivre la création et la mutualisation d'une base industrielle et technologique technologique de défense européenne. Considérant que l'OTAN reste aujourd'hui un frein réel et durable à la défense européenne, le groupe écologiste s'abstiendra. La parole est à M. Gilbert Roger, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes appelés ce matin à examiner le projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro.

des Balkans, se modernise et contribue à notre sécurité collective, notamment au travers de la lutte contre la corruption, le blanchiment et le crime organisé en vigueur sur son territoire. Son entrée dans l'OTAN lui permettra d'achever son processus de réformes démocratiques, institutionnelles et judiciaires en cours. Nous saluons cette démarche. Le Monténégro est un élément moteur de la coopération régionale dans les Balkans. Malgré sa taille modeste, il contribuera à la sécurité de l'Alliance en assurant le long de l'Adriatique un continuum un continuum géographique entre l'Albanie et la Croatie. Au niveau militaire, le pays a démontré son implication dans les missions de paix pilotées par l'Union européenne, notamment au Mali et en République centrafricaine.

été intégré au territoire russe ; il n'est donc pas dans la situation de l'Ukraine ou de la Géorgie. C'est la raison pour laquelle, si les autorités russes ont exprimé leur opposition à cet

de la politique dite « de la porte ouverte ». Aussi, ni la République de Macédoine, ni la Bosnie-Herzégovine, ni la Géorgie, ni, enfin, l'Ukraine ne sont en mesure de rejoindre l'OTAN dans les conditions actuelles. En effet, au-delà des difficultés que vivent ces différents États, l'évolution du contexte stratégique a conduit l'Alliance à se recentrer sur sa mission de défense collective, reléguant au second plan les questions d'élargissement. Enfin, l'adhésion du Monténégro à l'OTAN ne préjuge en rien des décisions que prendra, le moment venu, l'Union venu, l'Union européenne puisqu'il n'y a pas d'automaticité entre ces deux processus. Mes chers collègues, compte tenu de tous ces arguments, le groupe socialiste et républicain

je m'exprime sur le temps de parole du groupe Les Républicains, mais à titre personnel. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'excellent rapport réalisé par notre collègue, Xavier Pintat, sur un sujet rendu complexe par un contexte diplomatique et stratégique difficile. L'adhésion du Monténégro à l'OTAN peut paraître mineure au regard de la taille du pays et de son apport militaire et financier limité aux forces de l'Alliance atlantique. À titre d'exemple, seuls 1 850 hommes servent actuellement sous les drapeaux monténégrins. Sans vouloir sous-estimer les mérites de ses forces armées, on peut légitimement s'interroger sur la capacité réelle du Monténégro à contribuer à la sécurité de l'espace euro-atlantique, qui est pourtant, selon l'article 10 du traité de l'Atlantique Nord, l'un des critères devant présider à son élargissement. Cela dit, au-delà de l'intégration du Monténégro en elle-même, qui ne changera évidemment pas la face de l'OTAN, c'est bien le contexte dans lequel elle s'inscrit qui la rend problématique ; je fais bien sûr référence à la dégradation des relations entre les pays occidentaux et la Russie. À l'évidence, les agissements de Moscou en Ukraine exigeaient une réponse ferme et déterminée des Occidentaux, et tout particulièrement des Européens, car certaines lignes rouges ne sauraient être franchies sans conséquence.

Il n'est toutefois dans l'intérêt de personne de laisser perdurer des situations de tensions qui ne peuvent mener qu'à la surenchère et, finalement, à la montée des périls. La multiplication des démonstrations de force auxquelles nous assistons de la part de la Russie et de l'OTAN ces derniers mois en est le signe évident. On le sait, la Russie a une opposition de principe à tout élargissement de l'Alliance atlantique, qu'elle perçoit comme un encerclement portant directement atteinte Qu'il s'agisse ou non d'une surinterprétation des menaces qui pèsent véritablement sur elle, l'expansion de l'OTAN est donc indéniablement une source de crispations avec Moscou. Il ne s'agit bien évidemment pas de conférer à la Russie un quelconque droit de regard sur le processus d'élargissement de l'OTAN, qui appartient à ses États membres et à eux seuls, seuls, ni de souscrire à l'idée d'un partage de l'Europe en sphères d'influence. Cela dit, dans ce contexte tendu, les messages que nous envoyons sont particulièrement importants l'adhésion du Monténégro, guidée par des considérations plus politiques que stratégiques, constitue bien un message fort. Dans l'esprit de ses promoteurs, cette démarche est avant tout destinée à la région des Balkans occidentaux, dont le cheminement sur la voie de la stabilité doit encore être consolidé. on ne peut pas ignorer que ce n'est pas de cette manière qu'elle sera interprétée par la Russie. Bien que le Monténégro ne représente pas pour elle le même enjeu stratégique et symbolique que des États tels que l'Ukraine, la Géorgie ou encore la Serbie, les liens économiques et culturels, mais aussi militaires qui lient ces deux pays sont anciens et puissants. Même si les autorités russes ont déclaré qu'elles respecteraient la décision du Monténégro- c'est bien la moindre des choses, s'agissant du choix d'un État souverain

À un moment où nous devrions avant tout chercher le rétablissement de relations constructives, cette initiative me paraît donc particulièrement inopportune. Par ailleurs, cette adhésion doit également nous interpeller du point de vue des perspectives qu'elle dessine concernant un autre processus d'intégration, l'adhésion à l'Union européenne. En effet, l'adhésion à l'OTAN est généralement perçue comme un premier pas dans l'intégration à la communauté euro-atlantique, qui doit s'achever par une adhésion à l'Union européenne. Même s'il s'agit évidemment de deux processus totalement distincts juridiquement, force est de constater que les élargissements de l'OTAN menés depuis 1999 en Europe centrale et orientale ont tous débouché, sauf pour l'Albanie, sur une adhésion rapide à l'Union européenne. Il serait tout à fait irresponsable que cette logique perdure et que le Monténégro interprète son éventuelle accession à l'OTAN comme le signal d'une accélération à venir de ses négociations avec l'Union européenne. Je pense que, sur ce point, nous sommes d'accord, mes chers collègues. Disons-le d'emblée, nous ne pouvons donner aucune perspective d'adhésion au Monténégro, que ce soit à court ou à moyen terme. La capacité d'absorption de l'Union européenne est aujourd'hui saturée, même s'agissant d'un petit pays. L'Union doit concentrer ses efforts sur la redéfinition de son projet et de son fonctionnement avant de songer à s'élargir. Évitons de reproduire les erreurs des années 2000 Surtout, le Monténégro est encore loin d'être prêt à une telle adhésion, aux niveaux démocratique, institutionnel, économique ou judiciaire. S'il est vrai qu'il s'est engagé sur la voie des réformes pour renforcer l'État de droit et lutter contre la criminalité organisée et la corruption, les progrès enregistrés à ce jour n'empêchent pas qu'il soit toujours très éloigné des standards européens en la matière. Le fait qu'il soit soumis, depuis le début des négociations d'adhésion, en 2012, à une « nouvelle approche », reposant sur des exigences renforcées, en dit long sur la réalité de ce pays, qui n'a connu aucune alternance politique depuis plus de vingt-cinq ans et qui reste marqué par des soupçons de collusion avec des réseaux délictueux. Si la plus grande prudence doit prévaloir quant à la poursuite de la politique de la porte ouverte de l'OTAN, cela vaut donc encore davantage pour l'Union européenne. Je ne dis pas que le Monténégro ne pourra pas, un jour, rejoindre ces deux organisations, mais le contexte actuel, à la fois sur le plan international et sur le plan interne, devrait nous inciter à éviter toute précipitation. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous l'aurez compris, malgré toute la pertinence des analyses développées par notre rapporteur, je reste pour le moins circonspect

de loi de ratification. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Avant de mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi,

? Oui, monsieur le président.

C'est donc un jour important pour la lutte contre l'évasion fiscale, qui, tout au long du quinquennat, a été une priorité du Gouvernement. Le travail engagé depuis 2012 se poursuit aujourd'hui avec la ratification

et vous souvenez sans doute, en particulier, que la loi de finances pour 2016 a institué une obligation, pour les plus grandes entreprises, de déclarer à l'administration fiscale la répartition pays par pays des bénéfices et des principaux agrégats économiques comptables et fiscaux. Mais, pour être pleinement efficaces, ces déclarations doivent être échangées automatiquement entre les administrations fiscales, pour que chaque pays puisse avoir une vision globale de l'activité, notamment, des multinationales.

Je ne peux d'ailleurs que me réjouir que ce sujet essentiel transcende aujourd'hui les clivages partisans.

la France est favorable à un reporting public, dès lors qu'il sera la règle au sein de l'Union européenne. C'est la position que Michel Sapin

L'humilité commande de reconnaître que nous ne sommes pas encore parvenus au bout du chemin. Cela ne nous empêche pas de considérer que la France peut être fière de l'action qu'elle conduit en matière de lutte contre la fraude, tant au niveau national qu'au niveau international, pour au moins trois raisons. Premièrement, nous avons obtenu des résultats extrêmement intéressants, pour ne pas dire exceptionnels, dans la lutte contre la fraude fiscale. Ces résultats sont en progression constante. Ainsi, en 2015, l'administration fiscale a redressé 21,2 milliards d'euros de fraude, contre à peine 16 milliards d'euros, en moyenne, avant 2012.

Nous sommes parvenus à faire rentrer 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État : c'est plus que les budgets de la justice, de la culture et de l'aide au développement réunis

si ces résultats s'amplifient encore demain, ce sera grâce au rôle joué par la France à l'échelle internationale depuis 2012. Nous pouvons être fiers de la mise en place de l'échange automatique d'informations financières à compter de 2017, qui mettra fin au secret bancaire et fiscal entre 101 pays à l'échéance du 1 janvier 2018. Nous pouvons aussi être fiers de l'accord

On ne peut qu'espérer que, malgré l'évolution du contexte international, les engagements pris par chacun seront respectés. Je souhaite cependant rappeler que le mécanisme subsidiaire nous autorise à demander les informations aux filiales présentes sur notre territoire est implantée la maison mère ne nous les transmet pas. Une deuxième interrogation concerne l'utilisation que pourraient faire les autres pays de ces informations. l'accord prévoit des conditions strictes de réciprocité et de confidentialité. Bien entendu, nous veillerons particulièrement, avec l'ensemble de nos partenaires et avec l'OCDE, à ce que ces conditions soient respectées. Dans le cas contraire, nous suspendrions les échanges. Enfin, une troisième interrogation concerne la demande, légitime, d'une transparence plus large,

Doit-on s'arrêter là ? Bien sûr que non ! Un projet de directive est en cours de discussion à Bruxelles. La France souhaite qu'il soit adopté.

Si le secret fiscal et la liberté d'entreprendre nous interdisent une transparence totale- une transparence qui, du reste, ne serait pas forcément souhaitable -, il est important que chacun puisse avoir confiance dans l'action de notre administration. Nous devons rendre des comptes. Je comprends donc la démarche des auteurs de cet amendement. Au reste, je rappelle que, aux termes du paragraphe 3 de l'article 23 de la directive de 2011 sur l'assistance mutuelle, telle qu'elle a été modifiée par celle de 2016 sur l'échange automatique des déclarations pays par pays, nous allons devoir transmettre annuellement à la Commission européenne un questionnaire évaluant l'efficacité du dispositif. Je m'engage à ce que ces informations soient transmises à votre assemblée. Pour éviter de multiplier les rapports, je propose que ces informations soient présentées dans le rapport prévu à l'article 136 de la loi de finances pour 2011, qui porte sur les redressements

Je vous remercie

il s'agit des déclarations pays par pays auxquelles sont soumises les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 millions d'euros et qui sont transmises à l'administration fiscale. Ce dispositif a été introduit en France par anticipation au travers de la loi de finances pour 2016. L'objectif est de connaître les différentes filiales des groupes d'entreprises multinationales et de révéler d'éventuelles discordances de localisation entre les activités et leur imposition. La lecture des déclarations pays par pays à destination des administrations fiscales intervient donc en amont d'une éventuelle enquête approfondie, afin de déterminer les dossiers prioritaires. La déclaration pays par pays transmise à l'administration fiscale s'inscrit dans le cadre de l'action 13 du projet BEPS de l'OCDE, portant sur la documentation des prix de transfert. Afin de réduire les contraintes déclaratives pesant sur les entreprises, les États parties à la négociation sont convenus d'une déclaration unique auprès de l'administration fiscale du pays

entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du 29 octobre 2014, cet accord a été conclu sur le fondement de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de 1988.

Préférant conclure des accords bilatéraux, les États-Unis n'ont pas signé cet accord multilatéral. Cet accord organise les modalités de l'échange automatique des déclarations pays par pays sous condition de réciprocité, sous l'égide du secrétariat général de l'OCDE. Il précise également les conditions d'utilisation des données contenues dans la déclaration. En particulier, si elle permet une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert, la déclaration ne peut servir de base à des ajustements. Elle permet une analyse de risque préalable, afin de définir des priorités. Une enquête approfondie, conduisant notamment à analyser la documentation exhaustive des prix de transfert, doit ensuite être effectuée pour procéder à un éventuel ajustement. Par ailleurs, l'accord définit des procédures de consultation en cas de difficultés de mise en oeuvre, comme la non-transmission des déclarations par un État partie ou une utilisation inappropriée des données. des données. Une suspension temporaire ou définitive de l'échange automatique peut également être décidée par un État partie soit à l'égard d'un autre État partie, soit à l'égard de tous. Au-delà de ces précisions, j'approuve la conclusion rapide d'un accord équilibré qui permettra une application complète du mécanisme de déclaration pays par pays dès les premières déclarations sur l'exercice 2016, dix-huit mois après leur date de dépôt, soit à compter du second semestre de 2018.

avec les conventions fiscales bilatérales et les accords bilatéraux d'échange de renseignements fiscaux. Je souligne également que l'échange automatique des déclarations entre administrations fiscales des États membres de l'Union européenne est déjà prévu. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 25 mai 2016, la directive modifiant la directive de 2011 et prévoyant l'échange automatique des déclarations pays par pays entre administrations fiscales, la transposition des dispositions en droit national devant intervenir avant le 4 juin 2017. Chaque année, les États membres devront transmettre à la Commission européenne une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique des déclarations pays par pays, ainsi que les résultats pratiques obtenus.

Deuxièmement, un enjeu particulier réside dans la conclusion rapide d'accords bilatéraux avec les États qui n'ont pas signé le présent accord multilatéral et qui hébergent le siège de nombreux grands groupes d'entreprises internationales. Alors que le consensus né des négociations du projet BEPS, cristallisé dans les recommandations des rapports finaux d'octobre 2015, doit être transposé dans le droit, il convient que tous les États s'engagent. Je pense particulièrement aux États-Unis, qui ont introduit la déclaration pays par pays dans leur droit interne pour les exercices ouverts à compter du 30 juin 2016. Selon les informations qui m'ont été transmises, les États-Unis ont proposé à la France d'engager les négociations préalables à la conclusion d'un accord bilatéral d'échange. Mais cette matière relève des prérogatives du pouvoir exécutif : le renouvellement de l'administration américaine ne peut qu'accentuer nos incertitudes sur la position réelle des États-Unis sur ce dossier. Or leur implication est indispensable à deux titres : pour récupérer les données des groupes américains, mais aussi pour ne pas menacer le consensus né des négociations sur le Troisièmement, le projet BEPS prévoit une clause de réexamen en 2020. Grâce à une mise en oeuvre rapide, un premier retour d'expérience sera possible. Pour autant, le clivage qui existait, notamment, entre les pays hébergeant le siège de nombreux groupes et les autres, concernant les données à inclure dans la déclaration ou le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises y seront assujetties pourrait à nouveau apparaître.

Cet aspect est d'autant plus important que le multilatéralisme, s'il symbolise une volonté commune, conduit à inclure des États pour lesquels l'étanchéité des barrières entre services fiscaux et entreprises publiques doit être encore éprouvée.

Signé à Paris il y a tout juste un an, sous l'égide de l'OCDE- saluons au passage le dynamisme de cette organisation internationale -, cet accord rassemble une cinquantaine de pays unis par la volonté de lutter plus efficacement contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices vers les paradis fiscaux. Ce dispositif, déjà introduit dans le droit français par l'article 121 de la loi de finances pour 2016, oblige les entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dont le siège social est situé dans un pays donné à fournir à l'administration fiscale de ce pays une déclaration unique indiquant la répartition, pays par pays, de leurs bénéfices, mais aussi des principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux. Il prévoit également l'échange automatique de ces déclarations avec les administrations fiscales étrangères ayant adopté un dispositif équivalent.

L'accord respecte les principes de protection des données et de confidentialité, conformément à la convention internationale de 1988 relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ce qui exclut notamment le reporting public. Fruit d'un remarquable travail de négociation engagé en 2012 lors de la réunion du G20 de Los Cabos, cet accord va dans le bon sens. Il complète et généralise les accords bilatéraux conclus ces dernières années par la France avec certains pays, notamment les nouvelles conventions fiscales avec le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, Singapour et, dernièrement, la Colombie. Le RDSE

Ainsi, malgré le poids non négligeable des autres pays, notamment européens, l'absence de la première puissance mondiale réduit nécessairement la portée de l'accord, d'autant qu'il est permis de douter que la nouvelle administration américaine se montre particulièrement ouverte sur ce sujet Par ailleurs, rappelons que le reporting ne permet, en principe, à l'administration fiscale que de procéder à une « analyse de risque », et non à des redressements fiscaux, pour lesquels une enquête approfondie reste nécessaire.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

s'agit de la concrétisation juridique des engagements pris par les pays du G20 dans le cadre des travaux conduits par l'OCDE en vue d'apporter des solutions concrètes pour éliminer les failles permettant aujourd'hui à des sociétés d'organiser, biais de mécanismes d'optimisation permis par la combinaison de différentes législations fiscales, la « disparition » de leurs bénéfices ou le transfert artificiel de ces derniers vers des juridictions à faible fiscalité. Il s'agit d'une lutte perpétuelle qui devra être encore confortée.

est supérieur à 750 millions d'euros, de déclarer à l'administration fiscale la répartition, pays par pays, des bénéfices et principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que de communiquer des informations sur la localisation et l'activité des entités les constituant. L'article 223 C du code général des impôts prévoit également l'échange automatique de ces déclarations avec les administrations fiscales étrangères dotées d'un dispositif équivalent. En effet, une fois la capacité de collecte d'informations organisée, il faut mettre en place les conditions de l'échange entre les pays s'étant conformés à la recommandation n°13 de l'OCDE. Tel est l'objet de cet accord. Avec ce dispositif, l'efficacité du contrôle fiscal des grands groupes peut être renforcée par la mise à disposition d'une information pays par pays, couvrant une grande variété d'agrégats économiques. Le seuil retenu permettra de couvrir les 10 % d'entreprises multinationales réalisant environ 90 % du chiffre d'affaires mondial.

financière de 2008, les États membres du G20 ont pris conscience des coûts de l'évasion fiscale et ont érigé en priorité la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, afin d'améliorer la transparence du système financier international.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « les paradis fiscaux [ ...], c'est terminé », nous avait assuré, sans vraiment nous rassurer, le président Sarkozy le 23 septembre 2009.

concrétise une avancée majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale et le secret bancaire. Mis en oeuvre à l'échelle de cinquante États, la déclaration standardisée, pays par pays, et l'échange automatique des données entre administrations fiscales sont clairement de nature à entraver les transferts abusifs de bénéfices opérés par les grands groupes multinationaux à des fins d'optimisation fiscale dite « agressive

toutes les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui, y compris au coeur de l'Union européenne, ne sont pas abordées. Premièrement, si je me félicite, bien évidemment, de l'enquête lancée, vendredi dernier, par la médiatrice européenne sur les liens de M. Draghi avec l'industrie financière, je reste profondément atterré par notre tolérance collective aux conflits d'intérêts. Comment peut-on espérer lutter sérieusement contre l'évasion fiscale quand on porte à la présidence de la Commission européenne M. Jean-Claude Juncker, principal artisan du LuxLeaks, ou quand on autorise son prédécesseur, M. Barroso, à partir faire fructifier son carnet d'adresses chez Goldman Sachs ?

sont jugés sans recevoir le moindre soutien politique des gouvernements européens, alors même qu'ils ont grandement contribué, en dénonçant des pratiques désormais considérées illégales, à faire évoluer la législation.

Enfin, nous devons être très lucides sur la translation qui s'opère depuis quelques années : entre 2000 et 2015, parallèlement à la lutte contre les paradis fiscaux, le taux moyen d'imposition sur les sociétés au sein de l'OCDE est passé de 32 % à 25 %. Ainsi, en l'absence d'une véritable harmonisation à l'échelle européenne, c'est toujours le moins-disant fiscal qui est la norme. Néanmoins, parce que cet accord constitue bien évidemment une étape utile et nécessaire, le groupe écologiste votera en

En réponse à cette situation, et en application de l'accord BEPS, la loi de finances pour 2016 a institué une obligation, pour les plus grandes entreprises, de déclarer à l'administration fiscale la répartition, pays par pays, des bénéfices et des principaux agrégats économiques comptables et fiscaux.

de l'accord, je soulignerai que l'ensemble de ces mesures s'inscrit dans la droite ligne de l'action résolue menée par le Gouvernement depuis 2012 afin de lutter contre l'optimisation et l'évasion fiscales. Cette action ne cesse de faire la preuve de son efficacité : ainsi, en 2015, plus de 20 milliards d'euros ont été redressés, soit 5 milliards de plus qu'en 2012. Le volontarisme du Gouvernement en la matière s'illustre donc tout d'abord au niveau national depuis le début du quinquennat, plus de soixante-dix mesures de lutte contre la fraude fiscale ont été adoptées. Certaines d'entre elles visent tout particulièrement les fraudes reposant sur la dissimulation d'avoirs à l'étranger création du parquet national financier, à la taxation à hauteur de 60 % des avoirs détenus à l'étranger non déclarés dont la provenance n'est pas justifiée, ou encore à l'extension de six à dix ans des délais de reprise en matière d'impôt sur la fortune et de droits de succession au titre des biens ou droits non déclarés à l'étranger

La France s'est également investie dans la lutte contre l'érosion des bases fiscales. Elle travaille actuellement, avec près de quatre-vingt-dix autres pays, à la rédaction d'un instrument multilatéral qui puisse être adopté prochainement.

par des associations luttant de longue date contre ce fléau, telles que CCFD-Terre solidaire ou Oxfam, mais aussi par la Cour des comptes, qui a attesté d'une « impulsion politique nouvelle » faisant de la lutte contre la fraude fiscale « une priorité

Enfin, preuve que la politique mise en place par le Gouvernement fonctionne, les recettes liées aux redressements fiscaux ont progressé de 20 % en deux ans. Sur les plus de 20 milliards d'euros de redressements notifiés en 2015, les 12 milliards d'ores et déjà perçus représentent davantage que les budgets de la justice, de la culture et de l'aide et de l'aide au développement réunis, et autant que celui du ministère de l'intérieur ! Ces recettes supplémentaires liées à la lutte contre la fraude ont permis d'instaurer une baisse des impôts pour les classes moyennes et populaires.

sur le contenu de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 », notamment sur les articles concernant la publicité relative accordée au report des états comptables par pays d'implantation des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros. Cette mesure, déjà applicable au secteur bancaire et financier depuis la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, était notamment contestée au motif que, selon les députés et sénateurs requérants, « les les dispositions de l'article L. 225-102-4 du code de commerce méconnaissent la liberté d'entreprendre dès lors qu'elles contraignent les sociétés françaises à divulguer au public des informations de nature à révéler leur stratégie commerciale Par ailleurs, pour faire bonne mesure, les sénateurs requérants soutenaient également que « l'obligation ainsi instituée fait peser sur les sociétés qui y sont soumises une charge excessive contraire au principe d'égalité devant les charges publiques

objectif de valeur constitutionnelle, mais ils se sont tout de même permis une petite entorse au principe en indiquant, pour justifier la censure de l'article, que « l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale. Une telle obligation porte dès lors à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Cet accord constitue un pas important dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il est l'aboutissement d'un long processus de réflexion mené par l'OCDE, notamment depuis 2013, à la demande du G20. Au-delà de la lutte contre les paradis fiscaux et le secret bancaire, l'OCDE a souhaité étendre son action à certaines pratiques d'optimisation fiscale à travers le projet BEPS de lutte contre l'érosion des bases fiscales et le transfert des bénéfices. Ainsi, l'accord de janvier 2016 va permettre de rendre automatiques les échanges de déclarations, pays par pays, concernant les prix de transfert des grandes multinationales. Le principe du reporting pays par pays avait été adopté dans la loi du 30 décembre 2015 de finances pour 2016. L'obligation déclarative avait été créée, mais l'échange automatique des données, des données, sous condition de réciprocité, dépendait de l'adoption d'un accord international, qui fut signé quelques semaines plus tard, le 27 janvier Le présent projet de loi va permettre d'approuver cet accord et de mettre en oeuvre l'échange des déclarations pays par pays. Il faut noter que plusieurs tentatives des « frondeurs » de gauche visant à élargir l'assiette des entreprises concernées et à rendre publiques les informations ont échoué. échoué. L'article 137 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », a été censuré le 8 décembre dernier par le Conseil constitutionnel, au motif que la publicité des informations relatives à ces entreprises portait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Cet accord de janvier 2016 vise donc à lutter contre des pratiques abusives de certaines multinationales, liées aux prix de transfert. aux prix de transfert. Il s'agit des prix auxquels des entreprises d'un même groupe multinational, situées dans des États différents, se vendent des biens corporels, actifs incorporels ou services. Cette question est importante pour les administrations fiscales des pays concernés, car le transfert de bénéfices, à travers ces biens, actifs ou services, vers un pays à la fiscalité plus avantageuse peut permettre à des multinationales de diminuer de manière importante le montant de leur impôt sur les sociétés.

Pour vérifier ces prix, les administrations fiscales bénéficieront d'informations contenues dans les déclarations obligatoires transmises par les grandes multinationales, qu'elles s'échangeront automatiquement. Jusqu'à présent, elles n'avaient accès qu'aux informations concernant l'entité du groupe multinational présente sur leur territoire. L'accord de janvier 2016 a été signé par quarante-neuf pays, notamment par neuf des dix pays hébergeant le plus grand nombre de sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises mondiales.

retraçant, pour chacune des juridictions fiscales où elles exercent des activités, des éléments relatifs au chiffre d'affaires, au bénéfice ou à la perte avant impôts, aux impôts sur les bénéfices réellement acquittés ou dus pour l'année en cours, au capital social, aux bénéfices non distribués, au nombre d'employés, ainsi qu'aux actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. Afin de limiter la charge pesant sur les entreprises du groupe et de garantir davantage la confidentialité des données, une déclaration unique, pays par pays, est déposée, en principe dans la juridiction de résidence fiscale de la société mère. Elle fait ensuite l'objet d'une transmission automatique aux administrations fiscales des pays dans lesquels les filiales du groupe sont présentes, sous réserve de réciprocité. Cette déclaration ne concerne que les grandes entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires annuel consolidé dépasse 750 millions d'euros, afin que cette charge déclarative ne soit imposée qu'aux plus grandes entreprises, qui concentrent qui concentrent l'essentiel du chiffre d'affaires mondial. Cette obligation déclarative ne concernerait ainsi que 10 % des groupes d'entreprises multinationales, représentant environ 90 % du chiffre d'affaires agrégé des sociétés mondiales.

Sous réserve de quelques interrogations d'ordre technique, la commission des finances a adopté sans modification ce projet de loi, conformément à la position de son rapporteur Éric Doligé, dont je tiens à saluer la qualité du travail. En conséquence, conformément à la position que nous avons adoptée en commission, le groupe Les Républicains votera ce texte.

autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays. Mes chers